Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, M. le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l'article L.O. 320 du code électoral, Mme Brigitte Devesa est appelée à remplacer, en qualité de sénatrice des Bouches-du-Rhône, Patrick Boré, décédé le 5 juillet 2021. Son mandat a débuté le mardi 6 juillet 2021, à zéro heure.

et de santé au travail (SPST) de procéder à la numérisation des DMST, en conformité avec les référentiels d'interopérabilité et de sécurité du numérique en santé.

du code de la santé publique prévoit que tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.

Rappelons tout d'abord que ces données sont recueillies dans le respect de la plus stricte confidentialité. Les règles déontologiques applicables à ces professionnels interdisent logiquement qu'ils puissent tirer profit de leur activité en faisant le commerce de telles données. Pour rappel, le code de déontologie des médecins leur interdit déjà de tirer profit de leur intervention dans le cadre de leur activité professionnelle, d'en faire bénéficier des organismes au sein desquels ils exercent ou auxquels ils prêtent leur concours, voire de promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général. Enfin, la remontée des données des DMST vers la plateforme du Health Data Hub s'inscrit précisément dans une démarche d'intérêt général. En étant mises à disposition de la recherche scientifique, sous format anonymisé, elles doivent permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge de notre système de santé

interentreprises (SPSTI). Pour ce faire, les SPSTA doivent se doter de compétences identiques, y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, afin de répondre à l'ensemble des attentes et des besoins des employeurs et des salariés. Cette préoccupation

service de prévention et de santé au travail autonome peut être créé lorsque l'effectif de l'entreprise atteint au moins 500 salariés. Il est alors administré par l'employeur, sous le contrôle du Cet amendement tend à prévoir que les SPST autonomes se dotent de compétences pluridisciplinaires, y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP). En pratique, de nombreux SPSTA se sont déjà dotés d'une telle organisation. En outre, l'article 8 inséré par la commission introduit une possibilité pour les SPSTA de faire appel par convention aux compétences d'un SPSTI, notamment en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, ce qui répond au même objectif. De manière générale, ce sont toutefois les services autonomes qui ont tendance à capter la ressource médicale. L'exigence de pluridisciplinarité y est donc souvent moins cruciale. Par ailleurs,

L'agrément ne saurait donc en tenir compte. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, il s'agit d'un instrument dont la portée réelle est limitée et dont il ne faut pas trop attendre. Cependant, l'autorité administrative peut refuser la création du service, dont la petite taille pourrait constituer une fragilité

Ses participants ne suivant pas l'ensemble des salariés couverts par le service de santé, ils n'ont pas la capacité d'identifier l'ensemble des situations individuelles problématiques.

Cette cellule sera chargée de proposer des actions de sensibilisation, d'identifier les situations individuelles et de proposer, en lien avec l'employeur et le travailleur, un plan de retour ou de au travail. Afin de prévenir au mieux les risques de désinsertion professionnelle, il nous paraît indispensable de prendre le problème dans sa globalité en

C'est pourquoi nous souhaitons que la cellule créée ait également pour mission de proposer aux employeurs, en lien avec les salariés et leurs représentants, des plans de lutte contre les facteurs de risques psychosociaux, de désinsertion professionnelle, d'organisation pathogène du travail, de pathologie psychique relevant de l'épuisement professionnel, tels que le burn-out, de dépression et de suicide en lien avec le travail, d'accident et de pathologie du travail, ainsi que d'accident sur le trajet domicile-travail.

s'inscrit dans le même esprit que celui qui vient d'être présenté. Il s'agit d'expertiser les problèmes individuels des travailleurs, mais aussi les problèmes systémiques qui pourraient exister au sein des entreprises proposant des mauvaises conditions de travail susceptibles de constituer des facteurs de risques psychosociaux, de désinsertion professionnelle, de mauvaise organisation du travail, de stress, de burn-out, de dépression ou de suicide, d'accident sur le trajet du travail. Quel est l'avis de Ces deux amendements visent à compléter les missions de la cellule PDP mise en place par l'article 14 par des plans de lutte contre certains facteurs de risques psychosociaux, contre les pathologies psychiques, telles que le burn-out, ou encore contre les accidents de trajet. Il s'agit bien évidemment de sujets importants dont il faut tenir compte et sur lesquels les entreprises sont d'ailleurs loin d'être inactives. Toutefois, les plans de prévention, dont ces amendements chargent la cellule, vont bien au-delà de la prévention de la désinsertion professionnelle.

afin de laisser aux SPST les marges nécessaires pour mettre en place leur propre organisation, selon les spécificités de leur service, de leur territoire et des travailleurs suivis. Les expériences de terrain montrent que la prévention de la désinsertion

de la commission ? Si le texte issu de l'Assemblée nationale indique que la cellule PDP est pluridisciplinaire, il ne fixe toutefois aucune exigence quant à sa composition, laissant courir un risque de disparités entre territoires et entre secteurs professionnels. la commission a choisi de modifier l'article 14 afin de prévoir, d'une part, que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe des exigences minimales quant à la composition de la cellule, d'autre part, que l'animation et la coordination de cette cellule incombent à un médecin du travail.

Néanmoins, il ne paraît pas utile de préciser dans la loi toutes les possibilités d'organisation qui s'offrent aux SPSTI et qui sont très larges. En tant que rapporteur, je me dois de vous alerter sur cet écueil : des lois trop détaillées ferment davantage de portes qu'elles n'ouvrent de possibilités.

Alors que les entreprises de plus de vingt salariés ont l'obligation d'employer 6 % de travailleurs en situation de handicap, l'organisation des services de santé au travail est, dans certains cas, inadaptée pour répondre de manière réactive et efficace aux besoins de ces publics prioritaires. Afin de lever le frein au recrutement et à l'intégration des travailleurs en situation de handicap, nous proposons de leur réserver 6 % des créneaux de prise en charge. Pour adapter cette disposition aux particularités des services de santé au travail, ce taux est calculé au prorata de la part d'entreprises soumises à cette obligation.

en portage salarial seront bel et bien concernés par cette avancée que constitue la pratique de la télémédecine dans le cadre de la protection en santé au travail. On sait qu'il s'agit d'un moyen de dépistage important

dans le cadre de leur suivi de santé au travail. La possibilité du recours à la téléconsultation pour le suivi par la médecine du travail, introduite par l'article 15, s'entend pour l'ensemble des salariés qui sont suivis par le SPST

Que le travailleur soit suivi par le SPST autonome de l'entreprise de portage salarial ou par le SPSTI auquel elle est affiliée, à partir du moment où le SPST décide de recourir à un suivi par téléconsultation, il pourra le mettre en oeuvre

est à Mme Laurence Cohen. Si l'article 15 aborde les conditions des entretiens médicaux organisés par la médecine du travail, il ne s'agit pas là d'un progrès.

notamment sur la casse de la médecine du travail. Sans vouloir remettre en cause les qualités des internes en médecine du travail ou des infirmiers, nous réaffirmons que c'est au médecin du travail de conduire les visites médicales et non pas seulement de coordonner les équipes. Nous réaffirmons également que la santé des salariés nécessite des moyens ambitieux, c'est-à-dire des médecins du travail et non pas des solutions de repli pour cacher le manque d'effectifs. La démographie médicale dans cette spécialité a atteint un niveau critique. Le nombre de médecins exerçant actuellement suffit avec peine à couvrir les besoins de soins et de formation des futurs médecins du travail. Le seuil actuel de 5 000 médecins du travail est un minimum dangereux, quand on sait que leur moyenne d'âge est de 55 ans. Il en a d'ailleurs été pas mal question hier soir dans cet hémicycle. L'extinction progressive de la médecine du travail est une catastrophe. Elle entraîne une baisse de la qualité de la prévention, des complications évitables pour les expositions aux facteurs de pénibilité, le maintien de mauvais usages faute de conseil, mais, surtout, une difficulté de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles. Au-delà de la question démographique, c'est aussi une question politique garantir un suivi de médecine du travail de qualité, c'est garantir le droit des salariés, mais également tout l'édifice social de notre modèle de sécurité sociale tout au long de la vie. Ce modèle, depuis sa fondation par Ambroise Croizat, reste assis sur le travail. Tel est le sens de cet amendement.

du travailleur. En complément des modifications apportées par l'Assemblée nationale et des amendements adoptés par la commission pour renforcer la sécurité du recours aux téléconsultations, cet amendement, soutenu par la CFE-CGC, vise à poser

Dès lors, même si la pandémie a montré que le recours à la téléconsultation pouvait se révéler utile, nous tenons à réitérer que la présence physique du salarié et du médecin en rendez-vous médical doit rester le principe dans la très grande majorité des situations en temps ordinaire.

à même de juger si son rendez-vous médical peut se tenir à distance tout en respectant les règles de confidentialité. La téléconsultation est une bonne chose. Pour avoir présidé durant six ans un service de santé au travail,

ne saurait être considéré comme une norme et banalisé dans tout le secteur de la médecine du travail. De plus, à notre sens, les rencontres entre les salariés et le médecin du travail devraient se tenir en présentiel, dès que cela est possible, est possible, puisque la prévention et la sécurité des travailleurs passent par un entretien portant sur le corps, la posture et la présence physique et morale du travailleur. Nous savons que la téléconsultation ne permet pas un diagnostic

parole est à M. Éric Gold. La téléconsultation entre le médecin du travail et le salarié peut poser des problèmes de confidentialité et de discrétion lorsque le rendez-vous se déroule sur le temps de travail et sur le lieu de travail. Certaines configurations d'espace de travail, tels les, accentuent accentuent d'ailleurs ces difficultés. Aussi, pour ne pas pénaliser le salarié qui ne souhaiterait ou ne pourrait pas avoir recours à la téléconsultation, cet amendement vise à préciser que son refus n'emporte aucune conséquence.

M. Martin Lévrier. Téléconsultation, téléexpertise, télémédecine : autant de termes utilisés par tous, qui démontrent l'impact des nouvelles technologies sur la médecine moderne. Très utiles pour l'amélioration du parcours de soins, notamment auprès des populations résidant dans des déserts médicaux, ces outils ont prospéré pendant la pandémie. Pour autant, le Conseil d'État a estimé dans son avis sur cette proposition de loi que « la définition des actes de télémédecine est peu adaptée aux visites et examens réalisés dans le cadre de la médecine du travail L'article 15 prévoit d'autoriser le recours à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi des travailleurs. Tout outil permettant de renforcer la prévention et l'accompagnement de tous les travailleurs est bénéfique. Nous nous félicitons donc de cette mesure.

qui spécifie que le médecin traitant ou le professionnel médical consulté est choisi par le travailleur. En ce sens, il paraît opportun d'apporter ces modifications rédactionnelles de manière à apporter plus de souplesse dans l'usage des nouvelles technologies, avec comme objectif une meilleure prise en charge des travailleurs.

rectifié tendent à revenir sur la réforme de la santé au travail engagée dans la loi El Khomri de 2016, qui a remplacé la visite médicale d'embauche par une visite d'information et de prévention, sauf pour les salariés exposés à des risques particuliers. visite d'information et de prévention permet une prise en charge plus réactive par le service de santé au travail ; elle est assurée par un professionnel médical ou un infirmier. L'ANI sur la santé au travail n'est pas revenu sur cet équilibre.

Par ailleurs, notre commission a précisé les exigences de sécurité et de confidentialité qui seront applicables au recours à la téléconsultation, par analogie avec les exigences applicables à la télémédecine.

de l'article 15 est bien plus satisfaisant : l'opportunité de ce recours est laissée à l'appréciation du professionnel de santé, qui le proposera au travailleur ; le consentement de ce dernier conditionnera alors le recours à la téléconsultation. C'est pourquoi

d'une téléconsultation entre le professionnel de santé au travail et le travailleur associant le médecin traitant ou un spécialiste choisi par le travailleur, pour y substituer un échange à distance hors la présence du travailleur. Cette proposition exclut en réalité le travailleur du dialogue qui doit se développer entre le médecin du travail et le médecin traitant ou le médecin spécialiste. La configuration tripartite privilégiée par la commission est justement censée permettre la pleine participation du travailleur à la définition des solutions concertées entre ces professionnels pour garantir la coordination de son parcours de soins et sa conciliation avec sa vie professionnelle. Il convient de rappeler que le médecin traitant et d'autres médecins spécialistes sont désormais très largement incités à s'inscrire dans une démarche de collaboration avec les autres professionnels de santé qui suivent leurs patients, dans une logique de coordination des soins. Cela se fait notamment dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique,

à renverser le long processus de fragilisation de la médecine du travail, en rétablissant la visite médicale d'embauche transformée par la loi El Khomri en une simple visite d'information et de prévention, ce qui ne permet pas la prise en compte réelle de l'état de santé du salarié. cet amendement permettrait également de rétablir la capacité de cette visite à s'assurer de l'aptitude médicale du salarié à occuper son poste, également empêchée par la loi El Khomri. Ainsi, cet amendement tend à rendre au seul médecin du travail le pouvoir de mener cette visite médicale, qui ne pourrait pas être confiée à un autre professionnel de santé. Si l'on veut une prévention efficace, il semble logique qu'un véritable examen médical soit confié à un médecin. De plus, comme la périodicité des visites régulières est encadrée, cet amendement vise à la rendre annuelle pour tous les salariés et semestrielle pour les travailleurs de nuit. C'est pourquoi il serait souhaitable de l'adopter.

l'un des points de faiblesse du système de santé français. Alors, ne nous lamentons pas et n'ayons pas peur de la télémédecine ou de la téléconsultation ! Pourquoi

ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du salarié. La commission a transformé cette visite en un renforcement de la visite d'information et de prévention après l'âge de 45 ans. Cet article pose question, car sa plus-value n'est pas évidente. Dans un contexte de manque structurel de moyens alloués à la médecine du travail et de crise de la démographie des médecins du travail, on sait très

en médecine du travail, remis en cause par les réformes successives et par la passivité devant la démographie médicale, est à même de permettre une réelle prévention primaire et de prévenir la désinsertion professionnelle, dont l'âge n'est d'ailleurs pas le seul facteur.

si l'on estime que l'âge est un facteur important de désinsertion professionnelle, je vous propose d'acter qu'à partir d'un certain âge c'est au médecin du travail d'assurer des visites, afin d'être toujours en mesure de proposer à l'employeur des adaptations du poste de travail en lien avec la santé du salarié.

décisions politiques. Je rappelle que l'entretien de seconde partie de carrière est destiné à éviter toute pratique discriminatoire liée à l'âge dans les évolutions de carrière et devrait permettre au salarié d'anticiper la seconde partie de sa vie professionnelle par un examen de perspective de déroulement de carrière, en fonction de ses souhaits et, bien évidemment, au regard des possibilités de l'entreprise. Alors que les services de santé au travail peinent à remplir leur mission de suivi individuel des travailleurs, faute de moyens humains, cette mesure ouvre la voie à une remise en cause de l'obligation de visite quinquennale chez le médecin du travail. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Quel est l'avis de

La commission a réécrit cet article pour intégrer le contenu de cette visite au sein de la visite d'information et de prévention et de l'entretien professionnel pour les salariés de plus de 45 ans. Cette nouvelle rédaction permet de satisfaire l'objectif de l'ANI, qui est de mieux prévenir la désinsertion professionnelle en seconde partie de carrière sans créer de visite supplémentaire risquant de surcharger les services de santé au travail. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements

Ces amendements identiques tendent à rétablir l'article 16 dans sa rédaction initiale, qui crée une visite de mi-carrière à 45 ans. Bien entendu, la commission souscrit pleinement aux objectifs de cette visite, qui a été créée par l'ANI

elle manque aussi une partie de sa cible : les salariés dont les difficultés apparaissent après 45 ans, ceux qui ont des parcours hachés et qui ne seront pas en emploi à l'âge précis de 45 ans.

la commission a proposé d'intégrer le contenu de la visite de mi-carrière au cadre existant, c'est-à-dire à la visite d'information et de prévention et à l'entretien professionnel qui a lieu tous les six ans

Protéger les populations des maladies infectieuses est l'objectif des politiques de vaccination mises en place tout au long du XX siècle. Au titre de la lutte contre les épidémies, la vaccination est une composante de la politique de santé publique. Elle permet de combattre et d'éliminer les maladies infectieuses, potentiellement mortelles. On estime le nombre de vies ainsi sauvées Pour autant, le niveau de couverture vaccinale chez l'adulte est très insuffisant et inférieur aux objectifs de santé publique. Aussi, cet amendement vise à ce que la visite médicale de mi-carrière créée par l'article 16 soit l'occasion d'effectuer un bilan vaccinal.

Quel est l'avis de la commission ? Ces deux amendements tendent à préciser que, lors de la visite d'information et de prévention, le travailleur bénéficie d'une sensibilisation au risque d'exposition aux agents biologiques pathogènes et d'un bilan vaccinal.

de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de la sécurité sociale pour 2019, alors que le taux moyen de fréquence d'accidents du travail s'élevait à 33,5 %, ce chiffre atteignait 52,27 % pour les intérimaires.

Dans ce contexte, il importe de s'assurer que les intérimaires, mais également les professions indépendantes puissent profiter, comme les autres salariés, de la protection de la médecine du travail.

particulièrement menacés en raison de leurs conditions de travail souvent difficiles. Par cet amendement, nous tenons à nous assurer que les entreprises font le nécessaire pour protéger leurs intérimaires, en leur assurant une protection au travail à la hauteur de leurs conditions précaires de travail, qui les exposent à un risque bien plus important que la moyenne. Quel de la commission ? L'article 17 prévoit une possibilité de suivi par les SPST de l'entreprise utilisatrice des salariés intérimaires ou intervenant sur son site.

Dans le droit positif, le recours à un SPST n'est ouvert qu'aux travailleurs bénéficiant d'un contrat, c'est-à-dire aux personnes salariées. Pourtant, les travailleurs indépendants sont tout autant exposés aux risques liés à l'exercice d'une activité professionnelle. Que l'on soit indépendant dans le BTP, infirmier libéral ou assistant maternel à domicile, la pénibilité au travail est une réalité que personne ne saurait contester. Afin de lutter contre l'absence de recours au SPST, qui peut être justifié par de la négligence, par les emplois du temps chargés ou par la précarité financière et la recherche de contrats ou de clients, nous proposons une rédaction plus protectrice pour les publics concernés. En effet, nous savons tous que le non-recours au SPST participe aussi au diagnostic tardif d'une pathologie parfois grave. Nous vous proposons de miser davantage sur l'aspect préventif que sur le volet curatif, comme nous y invitent régulièrement les spécialistes de santé publique. En adoptant cet amendement, nous répondrons aussi à l'enjeu de la trop grande hétérogénéité en matière de santé au travail, qui a été dénoncée lors des auditions. Les deux

là aussi de garantir le principe de liberté des travailleurs indépendants d'être suivis ou non par un SPSTI.

de la commission ? L'article 17 précise que les travailleurs indépendants « peuvent » s'affilier au SPSTI de leur choix. Il s'agit donc bien d'une possibilité. L'amendement n° 149 vise à rendre cette affiliation obligatoire. Or ce n'est le souhait ni des partenaires sociaux ni de la commission. À titre personnel, j'y étais plutôt favorable, parce que je trouve que les travailleurs indépendants sont souvent bien seuls,

et la possibilité pour les travailleurs indépendants de renoncer à tout moment à leur affiliation. Nous avons déjà rejeté des amendements similaires en commission, car ils sont satisfaits par l'article 17, qui prévoit bien une possibilité d'affiliation. Par conséquent, la commission demande le retrait

Lubin. Il s'agit de permettre aux travailleurs des plateformes de bénéficier d'une protection élémentaire par un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Cette intention est satisfaite par les dispositions de l'article 17, qui ouvre la possibilité aux travailleurs indépendants de s'affilier aux SPSTI de leur choix. Pour l'instant, les travailleurs des plateformes sont juridiquement des travailleurs indépendants. Par conséquent, la

la proposition de loi prévoyait que les travailleurs indépendants pouvaient volontairement adhérer à un service de prévention et de santé au travail et, ainsi, bénéficier d'offres spécifiques à leur type d'activités.

La commission a prévu que le chef d'entreprise puisse bénéficier des services proposés par le SPSTI auquel son entreprise est affiliée sans hausse de cotisation, l'entreprise cotisant déjà pour ses salariés. Rappelons que les services des SPST sont facturés à l'entreprise, donc à l'employeur, et que le suivi facultatif du chef d'entreprise serait marginal pour des entreprises de taille certaine. L'amendement n° 165 tend à revenir sur la position de la commission, en supprimant l'absence de hausse de cotisations.

est à Mme le rapporteur. Compte tenu de la brièveté de leurs missions, d'une durée moyenne de quinze jours, les quelque trois millions de salariés intérimaires bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé très insuffisant et ne reçoivent presque aucune information de prévention sur les risques auxquels ils sont exposés, que ce soit par l'entreprise de travail temporaire ou par l'entreprise utilisatrice. Afin de compléter les dispositions prévues à l'article 17, qui ouvrent la possibilité aux SPST des entreprises utilisatrices d'assurer le suivi des intérimaires, cet amendement vise à renforcer les actions de prévention en santé au travail pour ces salariés.

Des actions de prévention sont déjà menées par les partenaires sociaux du secteur du travail temporaire, leur fonds d'action sociale. Pour une montée en charge de ces actions, il serait judicieux d'ouvrir, à titre expérimental, la possibilité que celles-ci soient réalisées par des professionnels de la santé au travail.

sur le fait que la suppression de l'article 17 posera un certain nombre de problèmes

l'article sur la mutualisation du suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès d'une pluralité d'employeurs,

et qui conduit les salariés remplissant les mêmes missions pour plusieurs employeurs à effectuer plusieurs visites médicales dans des services de santé au travail différents.

L'objectif de cette mutualisation est de rationaliser le système tel qu'il existe aujourd'hui, lequel conduit les salariés qui remplissent les mêmes missions pour plusieurs employeurs à effectuer plusieurs visites médicales dans des services de santé au travail différents.

conscients de la nécessité de renforcer la prévention et le suivi de l'état de santé de ces salariés, qui, compte tenu de leur situation, ne bénéficient pas d'une prise en charge satisfaisante. La commission a toutefois supprimé cet article pour deux raisons. part, il ne nous a pas semblé souhaitable que le législateur renvoie l'intégralité d'un dispositif à un décret, sans plus de précisions, au moins sur les grandes lignes de ce suivi spécifique. D'autre part, le Gouvernement a indiqué à l'Assemblée nationale qu'il ne serait certainement pas en mesure de prendre un décret pour définir ces modalités spécifiques.

Cela a été rappelé, l'obligation légale qui s'impose aux particuliers employeurs de s'occuper du suivi médical de leurs salariés est récente. Nous considérons évidemment qu'il s'agit d'une avancée, ces métiers étant

exercés au domicile soit des assistants maternels, soit des parents employeurs. Ces amendements, qu'il nous sera impossible d'examiner ici, mais sur lesquels je souhaite recueillir l'avis du Gouvernement, visaient à renvoyer à un accord de branche étendu

L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail [ ...]. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs

le Gouvernement considère que le suivi de la santé des salariés des particuliers employeurs est aujourd'hui très insuffisant. Ce secteur spécifique compte plus de 1,4 million de salariés et 3,4 millions d'employeurs.

Pour le Gouvernement, il est donc essentiel d'aboutir rapidement, en lien avec les acteurs du secteur, à un dispositif de prise en charge adapté. La commission des affaires sociales a adopté

Cette initiative permettra d'accélérer la mise en oeuvre de solutions véritablement opérationnelles et d'améliorer enfin le suivi de la santé au travail dans ce secteur. Le Gouvernement propose toutefois deux modifications à la rédaction de la commission afin de ne pas préjuger à ce stade de la forme de la contribution des employeurs qui sera mise en oeuvre

Compte tenu de la singularité de ce secteur, marqué par l'éclatement des employeurs et l'absence d'entreprise, il a semblé pertinent de prévoir la mutualisation de la gestion de la santé au travail par l'association

L'amendement n° 170 a pour objet d'apporter des précisions au dispositif adopté par la commission. Il tend à renvoyer à la négociation de branche l'ensemble des modalités de fixation de la cotisation, ce qui nous semble opportun. Il vise enfin à bien préciser que l'association paritaire qui agira pour le compte des particuliers employeurs désignera le ou les SPST compétents dans les territoires et conventionnera avec ces services.

de travailleurs visés par cet article ne doit pas faire l'objet d'une discrimination. Cette disposition a pour objectif de mettre fin à des situations inacceptables de discrimination systématique de la part de certains services de prévention et de santé au travail interentreprises. Elles se traduisent concrètement soit des refus nets de prise en charge, soit par des refus indirects, voire par des tarifs dissuasifs. Ces pratiques abusives doivent cesser avec cette réforme.

qu'un suivi adapté est ouvert aux « travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ». En outre, les itinérants peuvent avoir plusieurs statuts-

L'article 18 prévoit notamment une visite de reprise après un congé maternité ou une absence de longue durée liée à la maladie ou à un accident du travail. Ce rendez-vous de préreprise est présenté comme un outil pour l'employeur, le médecin-conseil et le service de santé au travail destiné à préparer au mieux le retour du salarié dans l'entreprise. Pour notre part, nous craignons que ce rendez-vous de liaison ne soit une source de confusion sur la nature des rapports entre les salariés

après une absence de longue durée et crée un rendez-vous dit de liaison entre l'employeur et le salarié. Bien que la commission ait ajouté, comme le recommandait le Conseil d'État dans son avis sur la proposition de loi,

En conséquence, nous proposons par cet amendement de supprimer la création de ce rendez-vous de liaison pendant la suspension du contrat de travail.

du salarié, au plus près de son collectif de travail. Elle doit intervenir en aval de la prévention primaire. Cet amendement de repli vise donc à préciser la nature du rendez-vous de préreprise afin de sécuriser les salariés.

ce qui nous semble très délicat pour le respect du secret médical. Il tend en outre à supprimer la possibilité pour l'employeur de solliciter le rendez-vous, ce qui ne nous semble pas souhaitable.

L'amendement n° 155 a pour objet de prévoir que le salarié doit être informé par l'employeur ou le SPST qu'il peut être accompagné, pendant le rendez-vous de liaison, d'un représentant syndical de son choix.

La visite de reprise est un élément fondamental pour agir en prévention de la désinsertion professionnelle d'un salarié. Elle est l'occasion d'échanger avec le salarié en cours d'arrêt de travail sur son état de santé, sa capacité à reprendre ou non et les outils pouvant accompagner sa reprise. Bien qu'elle soit prévue par le code du travail pour tout arrêt de plus de trois mois, cette visite est en réalité très peu réalisée.

les missions de prévention de la désinsertion professionnelle de la caisse de prévoyance sociale. Ainsi est garanti l'exercice effectif par la Caisse de Saint-Pierre-et-Miquelon de ses missions en matière de prévention de la désinsertion professionnelle- ou du maintien dans l'emploi, une expression que je préfère -, en lien avec les services de prévention et de santé au travail.

C'est dans cet esprit que l'Assemblée nationale a modifié la représentation des employeurs pour lui permettre d'être à l'image des entreprises couvertes. Il nous semble donc indispensable que cette disposition soit également appliquée à la représentation des salariés. Quel est l'avis de la commission ? Les signataires Quel est l'avis de la commission ? Les signataires de l'ANI n'ont pas entendu modifier les règles de désignation pour donner aux organisations représentatives un rôle dans une seule branche.

Haye. Depuis la création de l'article L. 4622-11 du code du travail, les collectivités territoriales ont pris l'habitude de faire appel au service de santé au travail pour assurer la surveillance médicale de leurs agents, afin de pallier les difficultés de recrutement des médecins de prévention. Celles-ci sont particulièrement présentes en Alsace, mais elles risquent de s'étendre aux autres régions. Cette proposition de loi, qui modifie la façon d'élire les représentants au conseil d'administration des services de santé, menace la présence des collectivités territoriales au sein de la gouvernance des services de prévention et santé au travail. travail. Elles ne pourraient plus alors veiller à la bonne prise en compte des particularités de la fonction publique, en particulier de la fonction publique territoriale. De même, elles ne pourraient plus participer à la discussion des évolutions de la santé au travail. Quel

3.1.4.4 prévoit ainsi que, « concernant les services de branches, les représentants des employeurs au conseil d'administration seront désignés par les organisations représentatives au niveau national et professionnel Il paraît donc essentiel de revenir sur les modifications adoptées en commission des affaires sociales afin d'assurer une juste représentation au sein du conseil d'administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises.

Leur gouvernance est actuellement assurée par un conseil d'administration et une commission de contrôle où siègent employeurs et salariés des entreprises adhérentes du territoire.

Le texte de la commission prévoit désormais la désignation des représentants des employeurs par les organisations patronales représentatives à l'échelon national et interprofessionnel. Nous proposons à travers cet amendement un levier pour améliorer le paritarisme dans les SPSTI, en ajoutant une règle d'alternance paritaire entre le collège des salariés et celui des employeurs

rappelle que la spécialisation en médecine du travail dure quatre ans -de contribuer au suivi de l'état de santé des travailleurs et travailleuses, en lien avec le médecin du travail. En prévoyant que des médecins de ville ayant suivi une formation, qui n'ont pas de connaissance de l'entreprise et qui ne peuvent pas se rendre sur le lieu de travail, contribuent au suivi des travailleurs, cet article dévalorise comme jamais, voire nie la spécificité de la médecine du travail, à l'heure où l'attractivité de cette spécialité devrait au contraire être soutenue.

Par ailleurs, la volonté de pallier le manque de médecins du travail par des médecins de ville est incompréhensible au regard des graves problèmes de démographie médicale observés dans de nombreux territoires, qui sont sur le point de devenir- ou sont déjà -des déserts médicaux. Je rappelle que le médecin de ville n'a pas accès à l'entreprise, alors que la proposition de loi rappelle par ailleurs dans d'autres articles l'importance du tiers-temps. Enfin, le système de « médecin collaborateur », qui permet à des médecins d'une autre spécialité qui se destinent à la médecine du travail d'être formés en théorie et en pratique au sein des services pendant deux ans, répond déjà de façon vertueuse à l'intérêt d'établir des passerelles entre la médecine de ville et la médecine du travail. Pour ces raisons, malgré les modifications apportées par la commission pour encadrer le recours aux médecins praticiens

une pénurie de médecins. Face au développement des déserts médicaux de généralistes, ce serait la double peine pour les salariés des territoires à la fois dépourvus de professionnels de la santé au travail et de généralistes.

Pourtant, au lieu de vous attaquer aux racines du problème en revalorisant les métiers et en améliorant l'attractivité des filières de médecins du travail, vous préférez bricoler avec les infirmiers et les généralistes des solutions tout de même assez bancales.

d'attirer de nouveaux étudiants non médecins. Il est nécessaire de renforcer les rangs des médecins du travail, spécialité à part qu'il faut par ailleurs rendre beaucoup plus attrayante. La parole

ne se limitent pas à la production de certificats de bonne santé ou d'aménagements de poste délivrés sans prendre aucune considération des réalités du terrain et de l'entreprise. La médecine du travail se situe au croisement d'une connaissance précise de l'état de santé du travailleur et des environnements des environnements et organisations de travail. Or, bien que soit prévue une formation en santé au travail du médecin « praticien correspondant », ce dernier ne pourra pas, comme le médecin du travail, se rendre sur le terrain et dans les entreprises pour saisir la réalité des conditions de travail du salarié et de l'environnement dans lequel il opère.

La nouvelle version de la proposition de loi prévoit que le médecin praticien correspondant devra conclure avec le service de prévention et de la santé au travail interentreprises un protocole de collaboration, signé à la fois par le directeur du SPSTI et le médecin du travail ayant autorité sur l'équipe pluridisciplinaire.

d'intégrer pleinement l'intervention du médecin praticien correspondant dans l'atteinte des objectifs du projet de service pluriannuel du SPST, en lui faisant partager à la fois l'approche populationnelle du service, adaptée aux spécificités des branches, secteurs d'activité et métiers suivis, et son approche par risque, selon les priorités fixées par le SPST en matière de prévention des risques. Par ailleurs, la commission a rappelé que le médecin praticien correspondant est appelé à être mobilisé quand les ressources médicales du SPST ne lui permettent pas d'assurer

? L'interdiction de cumul des fonctions de médecin traitant et de médecin praticien correspondant vise précisément à protéger le travailleur, en évitant que certaines informations liées à son état de santé, notamment en cas de pathologie chronique, viennent interférer dans sa vie professionnelle. Le cumul des fonctions

contre cette pénurie. Les législateurs qui se succèdent répètent à l'envi l'importance de la prévention dans la politique de santé au travail. Derrière les mots, les actes ne permettent pas d'enrayer la dégradation de la culture française de santé publique, en particulier dans la médecine du travail.

peu d'informations sur l'exercice de la médecine du travail durant la formation des étudiants en médecine ; des stages essentiellement réalisés à l'hôpital sous la direction de professionnels qui ne connaissent pas la médecine du travail ; aucune question relative à la santé au travail dans le concours de l'internat

Par ailleurs, la position de la commission est constante à l'égard des rapports : ils sont rarement remis dans les délais et ils sont assez peu suivis d'effets. L'avis est donc défavorable.

lors de laquelle les médecins du travail pourront délivrer à titre dérogatoire des arrêts de travail et prescrire des soins, examens ou produits de santé. Un médecin du travail est un médecin de plein exercice qui a le droit de prescrire, mais il le fait dans les limites de son rôle exclusivement préventif. Il peut notamment prescrire des examens complémentaires dans le cadre de l'article R. 4624-35 du code du travail. Bien que les médecins ne puissent pas cumuler plusieurs spécialités, ils peuvent avoir un exercice complémentaire dans le cadre de leur spécialité initiale. certains médecins du travail se sont déjà engagés dans une spécialité complémentaire, comme l'allergologie ou l'addictologie. Ils sont alors autorisés à prescrire si besoin dans le cadre de leur exercice complémentaire, mais cela doit rester dans un cadre préventif.

le ministre des solidarités et de la santé reconnaissait lui-même qu'en matière d'attractivité de la médecine du travail « un autre sujet réside peut-être dans la perte systématique de la capacité de prescrire des médecins du travail,

aux dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes. Il est pourtant essentiel que le temps clinique des SPSTI mis à disposition des entreprises et des salariés soit assuré. L'objet de cet amendement vise à permettre au médecin du travail d'assurer le suivi médical des salariés à risque, innovante de l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020,

M. Martin Lévrier. L'article 23 consacre dans la loi le statut d'infirmier de santé au travail et permet aux infirmiers en pratique avancée d'exercer au sein d'un service de prévention et de santé au travail. Les modifications adoptées par la commission des affaires sociales du Sénat, bien qu'énumérant les formations reconnues, apportent finalement une certaine rigidité à l'encadrement des critères permettant aux infirmiers et infirmières de voir leur formation reconnue. la rédaction restreint aux seules universités le champ de la formation. Or les instituts de formation en soins infirmiers disposent de toute l'expérience et des compétences nécessaires à l'enseignement des soins infirmiers en santé au travail. Il serait dommageable de ne pas permettre à ces instituts d'offrir cette formation spécifique. Notre amendement vise donc à offrir une plus grande latitude, tout en garantissant un niveau d'exigence de la formation qui sera défini par décret en Conseil d'État. L'amendement Mme Raymonde Poncet Monge. L'article 23 consacre dans la loi le statut d'infirmier de santé au travail et permet aux infirmiers en pratique avancée d'exercer au sein du service de prévention et de santé au travail. L'exercice L'exercice des infirmières et infirmiers en pratique avancée est encore trop peu reconnu- c'est un fait. Il apparaît urgent de valoriser comme il se doit le travail de ces professionnels. Pour ce faire, il est primordial d'y consacrer une formation universitaire spécifique et que celle-ci délivre un diplôme au grade de master.

Il va dans le sens des rapporteurs- permettre aux infirmiers et infirmières de santé au travail de suivre une formation sanctionnée par un diplôme universitaire. Il tend également à répondre à un manque dénoncé par le syndicat national des professionnels de la santé au travail, dont nous avons auditionné

Il n'y a pas de raison, selon nous, de traiter différemment le niveau de qualification attendu des infirmiers de santé au travail, compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées au titre du suivi individuel des travailleurs, de celui qui est reconnu aux infirmiers en pratique avancée.

En effet, tout comme les médecins du travail, les infirmiers et infirmières doivent pouvoir exercer en toute indépendance et à l'abri des pressions. Or, pour pouvoir exercer leurs missions, ils doivent être protégés du licenciement et des discriminations.

de santé au travail. L'article 23 prévoit la création d'un statut d'infirmier de santé au travail sans apporter de protection équivalente à celle dont bénéficie le médecin du travail.

c'est le médecin du travail qui dispose du statut de salarié protégé pour garantir son indépendance professionnelle vis-à-vis des entreprises adhérentes au SPST, parce qu'il est le seul et l'unique responsable des avis d'inaptitude et qu'il coordonne l'équipe pluridisciplinaire.

et les tâches qui pourront leur être déléguées. Les missions qui relèvent de la compétence spécifique du kinésithérapeute sont : l'évaluation et la prévention du risque physique ; la promotion de la santé de l'appareil locomoteur et le dépistage des troubles musculo-squelettiques avant le stade de la pathologie chronique ; la participation aux actions de promotion de l'activité physique ; la participation à la prévention de la désinsertion professionnelle, notamment pour les salariés présentant des restrictions physiques ou confrontés au risque physique ; la participation au plan de retour au travail pour ces mêmes salariés ; la possibilité, d'autant plus importante pour un effectif de professionnels qui sera réduit les premières années, de pratiquer des bilans ou des séances individuelles et collectives de conseil à distance grâce aux technologies de l'information et de la communication. Ces missions sont d'ores et déjà réalisées par les kinésithérapeutes depuis des années dans le cadre d'actions associatives, sur demande des employeurs. Cet amendement a donc pour objet de faciliter la collaboration entre les acteurs de la prévention et de la santé au travail dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires issues d'un même service. Quel est l'avis de ? La prise en compte des enjeux de santé au travail dans le parcours de formation des masseurs-kinésithérapeutes a effectivement été renforcée, notamment dans la prévention des affections de l'appareil locomoteur, du handicap et des troubles musculo-squelettiques. Toutefois, la présence des kinésithérapeutes au sein des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail reste encore très embryonnaire : selon l'association France Kiné Prévention, cinq masseurs-kinésithérapeutes exerceraient aujourd'hui dans des services de santé au travail. Du reste, des masseurs-kinésithérapeutes peuvent être non seulement recrutés par les services de santé au travail, mais aussi sollicités

d'un service de santé au travail. Cette formulation nous semble receler une ambiguïté, car elle pourrait laisser entendre que ces infirmiers devraient nécessairement être salariés d'un service interentreprises de santé au travail. C'est la raison pour laquelle nous vous soumettons cet amendement

en prenant appui sur la rédaction des alinéas 8 et 9 de l'article 23 adoptée en commission. Il s'agit ainsi de prévoir explicitement dans le code de la santé publique que, au titre de sa compétence en santé au travail, le ministère chargé du travail est également signataire de l'arrêté qui définit le référentiel de formation aujourd'hui fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de l'offre de formation. En l'état actuel de la rédaction, le ministère chargé du travail en est exclu ; c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

puisque cela suppose, en concertation avec les représentants des infirmiers et des établissements d'enseignement supérieur dispensant ces formations, de préciser les compétences cliniques et paracliniques qui devront être exigées de ces infirmiers. L'avis est donc défavorable.

En effet, les conventions internationales, notamment la convention du travail maritime et la convention n° 188 sur le travail dans la pêche, prévoient une visite médicale des marins au sein du SSGM tous les deux ans. Les infirmiers exerçant dans le SSGM ne sont donc pas amenés à recevoir les marins dans le cadre d'entretiens infirmiers, comme le code du travail le prévoit pour les entreprises terrestres. Ainsi, la formation spécifique en santé au travail prévue par l'article L. 4623-10 du code du travail créé par la présente proposition de loi n'apparaît pas nécessaire pour les infirmiers exerçant en SSGM. Le présent amendement vise donc à exclure les infirmiers travaillant au sein du SSGM de cette obligation de formation. Quel est l'avis de

La définition du contenu de cette formation requiert un temps de concertation et une adaptation des maquettes pédagogiques des formations proposées par les établissements d'enseignement supérieur les dispensant. En outre, afin de tenir compte de la recommandation du Conseil d'État dans son avis sur la proposition de loi, il est prévu une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des obligations de formation pour permettre aux infirmiers exerçant déjà au sein d'un SPST d'effectuer leur formation et d'obtenir le titre correspondant.

? Les professionnels de la santé bucco-dentaire collaborent déjà avec les services de santé au travail dans le cadre d'actions de prévention et de sensibilisation auprès de professionnels particulièrement exposés à des risques dans ce domaine, comme les boulangers-pâtissiers. Ce type de collaboration est bien calibré et adapté aux besoins des secteurs d'activité les plus pertinents. Il n'y a donc pas lieu de créer un statut de dentiste en santé au travail, dont il n'est pas sûr qu'il attire, en définitive, beaucoup de vocations. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.

L'article 24 consacre au niveau législatif la possibilité de délégation de tâches du médecin du travail à l'équipe pluridisciplinaire, étend son application et en prévoit les modalités spécifiques. L'intérêt de porter cette possibilité de délégation de tâches au niveau législatif n'est pas démontré ; en revanche, ces dispositions accentuent la démédicalisation, dans la la mesure où leur principal objectif- sinon le seul -est, comme d'autres dispositions de cette proposition de loi, de pallier la pénurie de médecins du travail en confiant leurs missions à d'autres professionnels : les infirmiers et infirmières en santé au travail ou les médecins correspondants que mentionne l'alinéa 6.

outre le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail et l'infirmier de santé au travail. Parmi ces auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, on dénombre bien entendu les masseurs-kinésithérapeutes et les ergothérapeutes, mais aussi les psychomotriciens.

Cette mesure est cohérente avec l'approfondissement de la pluridisciplinarité dans les services de prévention et de santé au travail souhaité par les partenaires sociaux dans le cadre de l'ANI du 9 décembre 2020 et poursuivi par toutes les réformes menées depuis 2011 sur les services de santé au travail. Elle permettra de mieux utiliser les ressources des services de santé au travail dans l'intérêt de la prévention dans les entreprises et des besoins des salariés. Ce choix, qui restera une faculté pour le médecin, sera en outre encadré par un décret en Conseil d'État, qui apportera toutes les garanties nécessaires.

C'est précisément de cette mission d'animation et de coordination que découle la possibilité pour le médecin du travail de déléguer, toujours sous sa responsabilité, d'autres tâches en lien avec le suivi médical des travailleurs, et c'est à ce titre qu'il dispose d'un statut protégé. La commission des affaires sociales est donc revenue

pluridisciplinaire de santé au travail pour la remplacer par un système de délégation de tâches. Les professionnels s'inquiètent des conséquences de cette disparition : l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire sont des composantes essentielles de l'indépendance des médecins du travail

L'ANI prévoit une organisation fonctionnelle en trois pôles qui constituent l'offre socle : le pôle prévention, celui du suivi de l'état de santé individuel des salariés et le pôle prévention de la désinsertion professionnelle. La responsabilité de l'organisation du service rendu aux adhérents doit relever de la direction du service et non du médecin du travail. C'est au directeur du SPSTI que revient le rôle d'organiser les missions de ses équipes. Cet amendement tend ainsi à inscrire l'ensemble des activités des médecins du travail, dans le respect de leur indépendance technique et dans le fonctionnement général du SPSTI défini au sein de leurs projets de service, pour que l'offre socle soit bien réalisée au bénéfice des employeurs et des salariés.

aux infirmiers et infirmières de santé au travail. La délégation de missions aux membres de l'équipe interdisciplinaire ne doit pas se faire au détriment du suivi du salarié comme du collectif de travail. comme du collectif de travail. Pour dire le lien entre santé et travail, le médecin doit pouvoir suivre régulièrement les salariés, en plus de son tiers-temps en entreprise. Or les visites médicales se sont espacées et raréfiées au fil des réformes, au point qu'un salarié peut ne jamais voir le médecin du travail pendant tout son parcours professionnel. Il convient donc de s'assurer, en complément des modifications bienvenues introduites par la commission, que les dispositions de l'article 24 n'aboutiront pas à confier aux infirmiers les visites médicales complexes.

Or l'équipe pluridisciplinaire est au coeur de la santé au travail et a accès aux professionnels et aux lieux de travail. Nous proposons donc, par cet amendement, qu'elle participe à un travail de sensibilisation sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre professionnel. implication permettrait d'améliorer et d'adapter les conditions de travail des personnes en situation de handicap sur le lieu de travail, mais aussi de lutter contre les préjugés et donc de créer une dynamique collective pour des embauches plus importantes. Cet amendement s'inscrit donc dans la suite logique de la création des référents handicap. Plus important sera le nombre de professionnels, sensibilisés et au travail sur le sujet, plus importante sera la part de personnes en situation de handicap insérées dans le marché du travail.

pour lui, de déléguer une partie de ses missions, comme c'est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui. L'avis est défavorable. L'amendement n° 186 rectifié, s'il était adopté, aurait pour effet de supprimer la condition de qualification pour bénéficier d'une délégation de tâches du médecin du travail. Or il est important que le médecin du travail délègue certaines de ses missions, sous réserve de la compétence du professionnel pour exercer cette mission. Par ailleurs, l'adoption de l'amendement aurait un effet contradictoire avec son objet : il tend à prévoir que les délégations de tâches ne pourront être réalisées qu'au profit des professionnels chargés du suivi de l'état de santé du travail ; or ces professionnels sont strictement définis par le premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail : il s'agit du collaborateur médecin, de l'interne en médecine du travail et de l'infirmier de santé au travail.

S'agissant de l'amendement n° 73, la loi prévoit déjà l'exclusivité de la réalisation de certaines visites par le médecin du travail, notamment l'examen médical d'aptitude après chaque embauche d'un travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. En outre, il est prévu qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail pourra déléguer une partie de ses missions, en tenant compte de la qualification du professionnel de santé délégué. Ce décret pourra exclure de la délégation de tâches certaines visites complexes dont la réalisation devra être réservée au médecin du travail. Par ailleurs, je rappelle que l'article 18 de la proposition de loi maintient bien la compétence exclusive du médecin du travail

Si les nombreuses défaillances de la politique de prévention en portent une part de responsabilité, il n'empêche qu'une partie de la solution pour retisser un lien de confiance entre les Français et la médecine passera également par la mise en place d'une véritable démocratie médicale. du patient ne peut plus se résumer à celui d'objet d'attention et de soins. Il doit être également reconnu comme un sujet dont les préférences doivent être écoutées et dont l'intervention individuelle ou collective doit peser sur les traitements et sur l'organisation des services de santé. Le patient, qui a acquis de solides connaissances de sa maladie au fil du temps, est devenu un acteur de l'éducation thérapeutique. Il s'implique auprès de malades souffrant de la même pathologie, mettant ainsi à leur service son expérience ; son savoir lui permet d'établir une relation de confiance avec les autres patients.

Cet amendement vise donc à modifier la composition du comité pour l'ouvrir aux associations de victimes du travail et de malades ainsi qu'aux syndicats. Leurs expériences et expertises sont importantes

Celles-ci doivent participer à la définition des politiques de santé au travail. Il est donc nécessaire de prévoir, au niveau législatif, que les organisations représentatives au niveau national et multiprofessionnel soient partie intégrante de ces instances. Cette précision se justifie plus encore au regard des missions dévolues au CNPST. Celui-ci sera donc en charge de définir l'offre socle des

sur un sujet aussi sensible que la santé et la sécurité au travail, les spécificités de multiples secteurs professionnels, notamment l'agriculture, forte de 1,2 million d'employés.

au comité national de prévention et de santé au travail, aux compétences étendues. La

créé par l'article 25, pour l'ouvrir aux associations de victimes du travail et de malades et de représentants d'usagers de la santé. Il nous semble en effet essentiel de renforcer la démocratie sanitaire en permettant à ces associations, fortes de leur expérience et de leur expertise, de participer et de faire des propositions. L'amendement Le handicap et sa prise en compte dans l'entreprise sont généralement traités comme un objet spécifique, indépendant de la santé au travail. Comme le souligne un rapport récent de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), l'activité professionnelle est en cause dans deux tiers des situations de handicap et la prévention en santé au travail constitue la première marche des politiques à mener en matière de handicap et d'emplois. Si l'enjeu commence à être perçu, les sphères d'intervention restent pourtant disjointes. Aussi, pour mettre fin à ce cloisonnement, cet amendement tend à intégrer les acteurs de la prise en charge du handicap au sein du comité national de prévention et de santé au travail. Il permettrait ainsi d'avancer sur les enjeux de la prise en compte du handicap dans les instances du dialogue social au sein de l'entreprise et du maintien en emploi lié au handicap au sein des dispositifs de prévention existants.

les partenaires sociaux n'ont pas prévu la participation à ce niveau-là. Le Gouvernement entend respecter cet équilibre et fait confiance aux partenaires sociaux et à leur capacité à améliorer la santé au travail,

alors que le texte prévoit de confier, au sein de l'instance, une voix par organisation syndicale et patronale. La présence de six organisations patronales contre cinq organisations syndicales représentatives entraîne une remise en cause de l'équilibre des parties. Les organisations syndicales ne sont pas opposées à la prise en compte de la diversité des organisations patronales, patronales, mais demandent à maintenir une parité de voix entre les différents représentants. Quel est l'avis de la commission

véritablement la représentation des organisations multiprofessionnelles.

M. Christian Bilhac. Par coordination avec un amendement défendu à l'article 25, le présent amendement vise à intégrer au sein des comités régionaux de prévention et de santé au travail, les acteurs de la prise en charge du handicap. handicapées (Agefiph), au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ou à Cap emploi. En effet, aujourd'hui, le handicap et sa prise en compte dans l'entreprise sont généralement traités comme un objet spécifique, indépendant de la santé au travail.

associatif régional. Il est déterminé à respecter le cadre juridique, comptable et financier, mais également le code des marchés publics. Il est en effet essentiel d'assurer la pérennité et la sécurité juridique et financière de cette agence et de son réseau qui ont montré toute leur utilité pendant la crise du covid-19 dans l'accompagnement des entreprises et des salariés. Cela implique une évolution profonde du réseau pour regrouper les agences régionales et l'Anact. cet amendement, en rétablissant l'article adopté par l'Assemblée nationale, permettra au Gouvernement d'agir par voie d'ordonnance pour assurer cette transformation. Cette évolution nécessite des transferts de biens, droits et obligations des associations régionales vers l'agence nationale. Ces dispositions appellent

se trouve entravé dans les faits par la dégradation des services de santé au travail et par l'insuffisance du nombre d'inspecteurs du travail, comme d'agents de la branche accidents du travail et maladies Sans représentant de ces services lors de leur réunion, les CSE perdent complètement leur sens. Le seuil requis pour la constitution d'un CSE et les stratégies de certains employeurs pour éviter le franchissement de ce seuil conduisent à ce que des pans entiers du monde du travail se trouvent exclus des dispositifs tendant à améliorer les conditions de travail. Les zones d'activités visées visées sont multiples, comme à Boulogne-sur-Mer, où la zone d'activités de Capécure, spécialisée dans la transformation des produits de la mer, rassemble 5 000 salariés répartis dans plus de 100 entreprises de taille diverses, sans compter un volant d'intérimaires mobilisables pendant les périodes de fêtes. Selon que l'on travaille pour Capitaine Capitaine Houat ou une PME, l'accès aux droits n'est pas le même pour tous, favorisant, par le jeu de la concurrence, le nivellement des droits par le bas. Dans cette zone, pourtant, les conditions de travail sont particulièrement pénibles : froid, humidité, risques de coupures et de mutilations, etc.

des représentants cités dans une instance unique. Ce qui est vrai pour Capécure l'est également pour les grandes zones commerciales, les zones d'activités autour de l'automobile ou de la verrerie. Il nous paraît donc important de créer des comités de site permettant de couvrir l'ensemble des à vous remercier

à un recours aux ordonnances. Du reste, je rappelle que l'article L. 1224-3 du code du travail prévoit déjà que « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ». En outre, ce regroupement n'a pas vocation à avoir un impact sur les missions de l'agence. De plus, son fonctionnement sur la base d'un réseau d'antennes régionales peut déjà être précisé par voie réglementaire. Mme Pénicaud l'avait rappelé,

on saisit mal, en pratique, comment seront regroupés les établissements sur la base d'activités de même nature. En effet, ces zones se caractérisent généralement par un tissu diversifié d'entreprises de tailles, mais aussi de secteurs d'activité très variables, confrontés à des enjeux de santé et de sécurité au travail très spécifiques. La commission a émis

Poncet Monge, sur l'article. L'article 28 concerne la formation en santé au travail des membres de la délégation du personnel du comité social d'entreprise. Puisque le CSE s'est vu attribuer des missions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, c'est l'occasion de rappeler que ce texte s'avère une occasion manquée de revenir sur les atteintes à la prévention en santé au travail, portées par plusieurs réformes antérieures. Parmi celles-ci,

cette opinion. Les CHSCT constituaient des institutions autonomes représentatives du personnel au sein des entreprises ou des administrations publiques. Leur objet était centré sur les questions de santé et de sécurité au travail, comme des conditions de travail, de façon spécifique et continue.

La suppression de cette instance de proximité a porté un coup inédit à la prévention en santé au travail et à l'analyse au plus près du travail réel et de ses conditions d'organisation. En effet, ces enjeux sont dilués au sein des CSE, avec des moyens en baisse très sensible, et seules quatre réunions annuelles ont l'obligation d'évoquer les sujets de santé, d'hygiène et de sécurité au travail. Le secteur de la prévention et de la santé au travail accuse encore le coup de la suppression de ce pilier de la prévention qui permettait l'expression des salariés sur leurs conditions concrètes de travail et sur les conséquences réelles des réorganisations en termes d'intensification du travail, de stress, voire de souffrance.

de la commission ? L'article 28 prévoit de rehausser la formation en santé, sécurité et conditions de travail des élus du personnel. Cette formation est uniformisée, quelle que soit la taille de l'entreprise, ce qui nous semble tout à fait bienvenu. Elle sera de cinq jours pour le premier mandat de membre de la délégation du personnel et pour tous les membres de la CSST des entreprises d'au moins 300 salariés. Elle sera de trois jours pour les autres membres en cas de renouvellement de mandat. Cette répartition, qui augmente déjà les durées de formation pour les entreprises de moins de 300 salariés, nous paraît adaptée et équilibrée- elle est même déjà

Au terme de l'examen de cette proposition de loi, notre sentiment général est une grande frustration. Nous n'avons pas discuté des véritables sujets de la santé au travail, comme la prévention primaire et le renforcement des droits des salariés.

Ma collègue Laurence Cohen l'a rappelé en début d'examen du texte lors d'un rappel au règlement, de nombreux amendements ont été déclarés irrecevables.

sans prise en charge financière des dépenses d'électricité et d'informatique, avec des dépressions liées à l'isolement ; je le rappelle, le télétravail

rien n'a été dit sur ce télétravail que des millions de travailleurs ont très mal vécu. Alors que la vague #MeToo a mis en avant la prévalence du harcèlement sexuel et sexiste en entreprise, rien n'a été dit, non plus Alors que, chaque jour, des médecins du travail partent à la retraite sans être remplacés, rien n'est fait pour favoriser les vocations de médecins. On a choisi de déléguer les tâches aux infirmiers et aux médecins généralistes, déjà débordés. Enfin, alors que la suppression des CHSCT a entraîné une perte énorme dans les entreprises, vous prétendez que leur transformation en commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique ne change rien. C'est complètement inexact.

met à mal ce type de réforme. Vous l'aurez compris, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera contre cette proposition de loi. explication de vote. Cette proposition de loi est décidément bien décevante. Nous regrettons qu'un texte qui portait l'ambition d'améliorer le suivi des travailleurs et la santé au travail n'apporte finalement que de la confusion et des risques.

Au total, il nous semble que les débats n'ont pas amélioré ce texte, tant s'en faut ! Les confusions créées nous semblent, au contraire, traduire une dégradation

travailler sur ce sujet, et de prendre un certain nombre de dispositions, notamment en ce qui concerne la prévention. Nous pensons également que le texte, tel qu'il a été travaillé par les rapporteurs et par la commission, est un texte de progrès.

amélioré par le travail des rapporteurs, que le groupe UC salue. Nous le voterons, comme nous l'avons dit dans la discussion générale. Le texte a été amélioré